chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je viens ici présenter ma proposition de loi pour la création d'un registre national des cancers. Avant tout, je tiens à remercier mon groupe, l'Union Centriste, d'avoir permis sa discussion, ainsi que tous mes collègues, sur toutes les travées du Sénat, qui ont largement soutenu ce texte. Je remercie également Mme la rapporteure, ma collègue Nadia Sollogoub, de son travail précis et argumenté, ainsi que la commission des affaires sociales, dont les apports ont modifié utilement le contenu du texte.

registre. Cet outil est déjà considéré comme indispensable par un très grand nombre d'acteurs pour améliorer et rendre plus efficace la lutte contre le cancer dans toutes ses dimensions.

sans la qualité du registre des cancers digestifs du Calvados et l'accès simple à ces données, ce travail n'aurait pas abouti. Nous avions alors mis en évidence une surincidence de cancers digestifs dans une population professionnellement exposée et exposée et une relation dose-effets entre la quantification de l'exposition à l'amiante et l'apparition d'un cancer digestif. Cela illustre parfaitement un fait : l'épidémiologie ne s'approche au plus près de la vérité scientifique

pour plusieurs raisons. Les constants progrès des diagnostics, la nécessité d'améliorer sans cesse le dépistage et la prévention, les besoins d'identifier les facteurs de risques émergents dans un environnement changeant où les expositions à des facteurs exogènes sont nombreuses et liées à l'évolution rapide de notre mode de vie,

Grâce à lui, j'ai pu assister à de nombreuses auditions qui ont constitué la base de son rapport et qui ont bien sûr alimenté ce travail législatif. C'est donc logiquement à l'issue d'un cheminement long et motivant que cette proposition de loi arrive aujourd'hui en examen au Sénat. s'est superposée une motivation supplémentaire. Parce que la révolution numérique permet aux données de santé de connaître un développement certain, et parce que l'intelligence artificielle laisse envisager des perspectives nouvelles, nul ne peut ignorer la nécessité d'un contrôle public ferme et exclusif du recueil

Ne soyons pas naïfs. Sur ces sujets, la avance, mais l'expertise et le contrôle humain dans un but de santé publique deviennent encore plus indispensables.

de mettre enfin un cadre à de nombreuses années de tergiversations pas toujours justifiées ni justifiables et de prendre la décision qui s'impose. Les outils et les compétences sont là.

N'étant ni médecin, ni chercheur, ni épidémiologiste, je n'ai pas osé formuler ma première réaction à cette proposition ; je pensais que c'était en place depuis longtemps. Et je suis certaine que nombre d'entre vous le pensaient également. Eh bien non ! Aujourd'hui, en France, les indicateurs de prévalence, d'incidence, de mortalité et de survie du cancer dont nous disposons sont des estimations au titre de l'année 2018, extrapolées à partir de 24 % de la population. Tout d'abord, je dois rappeler que les registres des cancers sont des outils, des recueils de données individuelles nominatives. Concrètement, les personnels des registres, des techniciens spécialement formés, vont chercher les informations nécessaires auprès de différentes sources- laboratoires d'anatomopathologie, laboratoires de biologie, établissements de santé, publics et privés, assurance maladie, réseaux de cancérologie, centres régionaux de dépistage du cancer -, afin d'assurer l'exhaustivité du repérage des patients. Ils consultent également les dossiers médicaux dans les établissements pour recueillir tous les items indispensables à la description du patient et de sa pathologie. La composante humaine de l'investigation permet la compréhension du parcours de soins dans sa globalité. De l'avis général des spécialistes que nous avons auditionnés, le travail effectué sur le terrain conditionne la qualité des données. Aujourd'hui, un parcours de soins est haché, et il existe beaucoup de données de santé chez le généraliste, chez le pharmacien, à l'hôpital ... Aller chercher ces données suppose des recherches et prend du temps. Les registres des cancers ont été créés progressivement depuis les années 1970. Il existe actuellement dix-neuf registres généraux couvrant vingt-quatre départements, dont cinq ultramarins, douze registres spécialisés pour certains types de cancers, deux registres nationaux pour les cancers des enfants et des adolescents, et deux registres nationaux pour les mésothéliomes pleuraux et les tumeurs rares du péritoine. Il s'agit d'outils très complets, dont l'unité d'enregistrement est l'individu. Les modalités de gouvernance et de financement du système sont cependant complexes. La base commune des registres, qui sont regroupés depuis 1995 au sein du réseau Francim, est hébergée par le service de biostatistiques des Hospices civils de Lyon, et gérée conjointement par l'INCa et Santé publique France, qui sont aussi les premiers financeurs de registres, à hauteur des deux tiers. Souhaitons-nous soutenir dans nos politiques publiques la montée en puissance de cet outil potentiellement très puissant, qui permet de mieux connaître le cancer, et donc de le combattre ? Je rappelle que l'on parle de la première cause de décès chez l'homme, et de la deuxième chez la femme. Si oui, il faut d'abord écouter les opérateurs et utilisateurs de ces données, qui nous demandent plus de souplesse dans leur interopérabilité et leur accès. D'autres bases de données, tel le Système national des données de santé (SNDS), regroupant des données de consommation de soins dans un objectif économique, mais couvrant l'ensemble du territoire français, doivent pouvoir être croisées le plus simplement possible avec celles des registres. de même, par exemple, pour les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). Que ce soit pour les expositions environnementales, les expositions professionnelles ou les trajectoires de soins, le croisement des bases de données est indispensable. Or il est actuellement réalisé de manière probabiliste dans la majorité des travaux.

complète dans la durée. Dans le prolongement, il faudrait, par voie réglementaire également, autoriser aux registres l'accès aux certificats de décès nominatifs et aux données de mortalité en général. en général. Cette proposition législative vise à doter la France, comme beaucoup de nos voisins européens, d'un outil harmonisé, global et exhaustif, couvrant l'ensemble du territoire national. Évidemment, cette construction se fera dans le respect des outils actuellement en place, qui sont solides et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Une forte demande émane du monde associatif, des patients en général, tout autant que de scientifiques et de responsables administratifs. Le rapport de 2017 de Bégaud, Polton et Von Lennep encourageait à constituer des registres nationaux en cancérologie pour certaines molécules, afin de donner tout leur potentiel aux données en vie réelle, ce qui fait toute la différence avec les recherches sur un échantillon de patients sélectionnés. En 2020, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) relevait, en évaluant le troisième plan cancer, que « des données à une échelle géographique plus fine sont nécessaires En 2021, le Haut Conseil de la santé publique plaidait pour une meilleure homogénéisation des données et la création d'un dispositif national de détection des signaux faibles. nationale de médecine, enfin, a appelé plus clairement en 2021 à la création d'un registre national des cancers, accompagné d'un mécanisme de déclaration obligatoire de la maladie, afin d'accélérer les remontées d'informations nécessaires à l'exercice d'une mission de surveillance sanitaire élargie. J'ai été maire d'une commune située à deux kilomètres d'une centrale nucléaire, et je vous confirme la forte demande des populations pour un maillage territorial fin, permettant une connaissance précise, particulièrement à proximité des sites sensibles ou pollués, comme l'a souligné notre collègue Émilienne Poumirol. Prévenir plutôt que guérir, mais aussi tordre le cou aux rimeurs, éviter les théories du complot. On sait qu'elles fusent vite et qu'elles sont difficilement contrôlables ... Si la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui fait suite à de multiples préconisations, y compris scientifiques, il faut dire que certains ont également exprimé des réserves sur la balance coût-efficacité de l'opération. Je note à ce sujet, d'une façon générale, l'extrême inquiétude du monde de la recherche, déjà entendue lors d'un colloque à l'Académie nationale de médecine, quant à la difficulté d'accéder aux crédits qui leur sont consacrés, souvent dilués dans des budgets globaux, peu lisibles, difficiles à sanctuariser.

alors que le nombre de cancers augmente. On peut comprendre cette inquiétude devant la fragilité des financements, qui motive certaines réserves, en particulier celles de l'INCa, mais il serait tellement dommage que le monde de la recherche s'autocensure Faire le choix de conserver des données parcellaires alors qu'il faut une information la plus précise possible pour planifier l'offre de soins serait par ailleurs difficilement compréhensible. Certes, tout cela a un coût Comme je vous l'exposais en propos liminaire, les opérateurs des registres passent beaucoup de temps à rassembler des données. On nous a même dit que les chercheurs eux-mêmes passaient un temps énorme à saisir des données, voire à chercher des financements, temps qui n'est pas consacré aux travaux de recherche. La généralisation d'une base de données nationale et la mise en commun de nombreuses informations permettront d'optimiser les opérations de saisie et rendront du temps à la recherche. Elles permettront également d'éviter les doublons et les manquants, d'avoir une veille sanitaire plus large et de régler le problème du suivi des patients dans leur mobilité géographique : ceux-ci seront suivis dans leur environnement et leur contexte. L'enregistrement systématique en continu de toutes les données permettra enfin de réduire les délais de production des rapports. Et n'oublions pas non plus, mes chers collègues, que les données de santé ont un coût, mais également un prix Si les industriels ne trouvent pas en France les données sur les cancers dont ils ont besoin pour mettre au point leurs traitements, ils iront les acheter ailleurs : en Allemagne, qui est en train de se doter d'un registre national, ou au Royaume-Uni, qui en dispose déjà. C'est un vrai enjeu de compétitivité mondiale et de souveraineté de la France. La recherche avance chaque jour. Le niveau de connaissance de chaque pathologie s'affine. On ne peut plus parler désormais « du cancer » : il faut parler « des cancers », que l'on individualise de mieux en mieux. En poussant le raisonnement, on pourrait presque considérer que chaque cancer sera bientôt un cancer rare, d'où l'intérêt des cohortes les plus larges possible, internationales ou au moins européennes, qui seront forcément plus pertinentes que les extrapolations ou les échantillons. Après que le plan Cancer a créé en France l'INCa, qui est un modèle envié, il y a une vraie logique à mettre désormais entre ses mains un registre national des cancers, qui concentrera des données fiables, exploitables et, surtout, extrêmement utiles.

ces mots du président d'honneur de la Ligue contre le cancer, le très regretté professeur Axel Kahn, transparaît ce qui nous rassemble et nous anime : nous engager, nous investir et innover, pour avancer chaque jour dans l'amélioration des connaissances scientifiques en oncologie, qui permettent de toujours mieux traiter et mieux accompagner les patients souffrant d'un cancer. Je sais que c'est l'objectif qui a présidé à l'élaboration de cette proposition de loi. je tiens à saluer l'engagement qui est le vôtre, madame la rapporteure, en tant que représentante politique et en tant que médecin, pour faire avancer cette cause importante, ainsi que le vôtre, madame Sonia de La Provôté, qui l'avez rappelé dans votre préambule. La cause est importante et nous concerne tous. Près de 4 millions de nos concitoyens vivent aujourd'hui, à différents degrés, avec le cancer. Derrière les diagnostics, toujours difficiles, il y a des individus qui se battent. Il y a des vies, des familles et des projets que l'on peut reconstruire. Oui, le cancer tue ; le cancer laisse souvent des fardeaux de séquelles. Mais, aujourd'hui, grâce aux progrès de la science, on peut guérir du cancer. Grâce aux avancées de la médecine, les traitements sont de plus en plus ambulatoires, de moins en moins aliénants et plus faciles à supporter : on vit mieux avec le cancer. Dépistage, prévention, prises en charge innovantes, nouvelles thérapies ... sont autant d'armes contre le cancer, qui font que les chances de guérison des malades progressent de jour en jour. Au XXI siècle, nous touchons réellement et résolument du doigt l'espoir de vaincre cette maladie. À la racine de tous ces progrès, de tous ces espoirs et de toutes ces avancées, il y a toujours la recherche scientifique, notamment la collecte et l'analyse de données, qui nous permettent de progresser, chaque jour, dans l'évaluation des facteurs de risque du cancer ou dans la classification des tumeurs. En effet, que ce soit en épidémiologie, bio-informatique ou biostatistique, la data est une clé majeure pour mieux comprendre les différents cancers et leurs spécificités. En effet, le terme « cancer » recouvre plus d'une centaine de maladies différentes, sans compter un grand nombre de sous-catégories. Aussi, c'est une priorité forte du ministère de la santé et de la prévention que de se donner les moyens d'observer et de suivre, de manière exhaustive et approfondie, la prévalence, les déterminants et les évolutions des cancers, pour agir de la manière la plus anticipée et la plus ciblée possible sur la maladie. En matière de données de santé, il faut souligner combien notre pays est avancé et dispose d'atouts considérables. Notre SNDS, en particulier, est un ensemble unique au monde par sa richesse et son exhaustivité. Il est composé de toute la base médico-administrative de l'assurance maladie, mais aussi du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), ainsi que du registre des causes de décès. Le cancer est une maladie qui nécessite un suivi et des soins coûteux prolongés. À ce titre, tous les patients atteints sont naturellement, de droit et automatiquement, considérés comme relevant du régime de l'affection de longue durée (ALD), qui leur permet de bénéficier de soins pris en charge à 100 % par l'assurance maladie. Ainsi, mesdames, messieurs les sénateurs, les données relatives au traitement de chacun des patients pris en charge en France pour un cancer sont déjà répertoriées dans notre système national des données de santé. sans compter la multiplicité des initiatives complémentaires. Je pense aux registres spécialisés, pour les cancers digestifs ou les cancers pédiatriques, par exemple, ou encore à l'Onco Data Hub, piloté par Unicancer. La mise en place de Mon espace santé, le carnet de santé numérique, créé pour déjà plus de 60 millions de nos concitoyens, ouvre également de nouvelles perspectives pour une vision, qualitative et quantitative, toujours plus exhaustive de l'état de santé de la population et de son évolution, en particulier concernant le cancer. Vous le voyez, la croissance des données émises, stockées, utilisées et échangées chaque jour par les établissements, administrations, laboratoires et professionnels de santé est exponentielle. C'est pourquoi, aujourd'hui, le débat n'est pas tant de constituer une base de données nationale des cancers, qui, je le répète, existe, et s'enrichit en temps réel. L'enjeu est de mettre cette ressource précieuse au service des progrès de la recherche et de répondre au défi d'avenir que constitue le traitement algorithmique des données de santé. C'est tout l'objet de la mise en place, depuis 2019, de la Plateforme des données de santé. Cette infrastructure numérique innovante nous permet de faciliter le partage et, surtout, l'analyse croisée des données de santé, issues de sources variées, et, en premier lieu, de la base anonymisée du SNDS. La dynamique actuelle de La dynamique actuelle de déploiement d'entrepôts de données de santé hospitalières vient soutenir cette démarche. Avec 40 millions d'euros de financements dédiés, issus de la stratégie d'accélération de la santé numérique du plan France 2030, sélectionnés. Ces lauréats, pleins de potentiel, constituent la première pierre d'un vaste réseau national interopérable de production partagée et de partage fluide de données hospitalières que nous voulons, à terme, constituer. Ces données hospitalières sont particulièrement profitables à la recherche en oncologie. Elles viennent utilement compléter les informations administratives de l'assurance maladie d'informations cliniques de « vie réelle Ces données de « vie réelle » sont les plus utiles, les plus pertinentes et les plus intéressantes. C'est pourquoi nous continuons de resserrer le maillage des hôpitaux équipés pour le traitement de leurs données. La seconde vague de l'appel à projets d'entrepôts hospitaliers a ainsi bénéficié d'une enveloppe supplémentaire de 25 millions d'euros. Il faut bien garder en tête que la valeur de toutes ces données de santé n'est pas intrinsèque. La valeur de la donnée est définie par son utilisation, et non par sa nature, par le service rendu pour l'utilisateur, et les progrès qu'elle permet. Elle est proportionnelle à la connaissance intégrée et se détermine par le niveau de partage, la qualité et la quantité des échanges et des connexions qu'il est possible d'établir entre les différentes sources de données. Ainsi, il s'agit tout autant d'explorer toutes les possibilités d'usage et de valorisation de ces données que de développer encore de nouveaux outils technologiques qui auront la capacité de décupler leurs facultés, par exemple en observant différentes échelles simultanément et en multipliant les croisements d'informations. C'est ce à quoi s'attachent aujourd'hui nos organismes spécialisés dans la lutte contre le cancer, comme l'INCa, institution à laquelle je veux rendre hommage et dont je salue l'expertise sanitaire et scientifique des membres. C'est également l'un des objectifs majeurs poursuivis lorsque nous déployons des efforts inédits pour mettre en place et développer dans notre pays les structures de pointe que sont les instituts Le premier biocluster, inauguré au mois de février dernier, le Paris-Saclay Cancer Cluster, est d'ailleurs centré autour de l'enjeu qui nous préoccupe aujourd'hui, comme le reflet de l'importance prioritaire que le Gouvernement attache à cette question. Je voudrais aussi mentionner combien il est important, pour avancer dans la connaissance du cancer, d'adopter une vision globale. Les données concernant la maladie doivent être croisées entre elles, mais aussi mises en perspective avec toute la richesse qu'offre notre système national, et même au-delà. La recherche contre le cancer ne pourra que bénéficier d'un meilleur partage international des informations administratives, cliniques et statistiques. Sur cette question aussi, la France fait figure de leader. La présence du Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Lyon, où sont mises à disposition des chercheurs les bases de données mondiales de référence en oncologie, nous permet d'enrichir encore notre panel scientifique en la matière. Vous l'aurez compris, si je soutiens tout à fait la démarche transpartisane à l'origine du texte que nous examinons, il me semble bel et bien qu'en 2023, l'heure n'est plus à la constitution de registres Nous disposons aujourd'hui d'une ressource formidable, exhaustive et immense en matière de données de santé, et particulièrement en oncologie. Le défi du XXI siècle est, je le crois, de concentrer nos efforts à en explorer les possibilités. J'entends néanmoins vos arguments, qui témoignent de l'importance que vous accordez à cet enjeu prioritaire. C'est pourquoi, malgré les réserves exprimées sur l'opérationnalité de la mesure et, surtout, conscient que la lutte contre le cancer doit mobiliser les énergies et les bonnes volontés, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat sur cette proposition de loi, en soulignant que, si la navette devait se poursuivre, le texte nécessitera encore un travail collectif soutenu. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi de ma collègue du groupe Union Centriste Sonia de la Provôté, qui vise à mettre en place un registre national général des cancers, géré par l'Institut national du cancer. Cette proposition de loi a été cosignée par la quasi-totalité des membres de notre groupe et, au-delà, par une centaine de membres de la Haute Assemblée au total, ce qui démontre l'intérêt et la pertinence de ce texte. Cela a été souligné, mais je tiens à le rappeler : le cancer est la première cause de mortalité pour les hommes et la deuxième pour les femmes. Le nombre de décès dus au cancer est estimé à plus de 150 000 par an. La lutte contre cette maladie apparaît donc comme une priorité, et ce registre national des cancers comme un outil essentiel en cancérologie. La création de ce registre national fait consensus sur son utilité et sa pertinence, mais quelques réserves ont été émises quant à son coût financier par l'Institut national du cancer, qui sera chargé de sa gestion. Or il nous semble que le coût généré représentera, sur le long terme, une économie d'échelle et un investissement pour la recherche et la prévention. nationale de médecine préconise de garantir la pérennité de son financement en optimisant l'utilisation des finances publiques et en mobilisant des fonds dédiés au programme national du numérique en santé. Madame la ministre, quelles mesures entendez-vous prendre sur le sujet ? Pouvez-vous rassurer l'INCa en garantissant que, si cette proposition de loi devenait loi, une augmentation de ses crédits serait prévue en la prise en charge actuelle des cancers s'élève, en 2020, à 5,9 milliards d'euros de dépenses hospitalières, liées au diagnostic, au traitement ou au suivi des personnes malades. Un registre national serait un outil déterminant au service d'une priorité majeure pour la santé publique une véritable politique de prévention d'une maladie dont l'incidence a augmenté, en trente ans, de 65 % chez les hommes et de 93 % chez les femmes. Il existe actuellement 33 registres, 19 registres généraux, couvrant 24 départements, et 14 registres spécialisés dans des cancers localisés dans des organes spécifiques. Au total, ils ne couvrent que 22 % de la population française. C'est donc par extrapolation que les données sont établies. Madame la ministre, vous ne me contredirez pas si je dis que le corps humain n'est pas une formule mathématique. Ce sont bien les effets de l'environnement et les mutations induites qui nous ont fait passer de Luca, dernier ancêtre commun universel, à. En matière de santé, chaque individu possède des spécificités et nos territoires nous exposent de manière différente. La recherche en santé ne peut donc pas se satisfaire de l'extrapolation et de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, notre rapporteur, que je salue, a souligné la sous-exploitation du potentiel des registres : le panorama fourni par leurs données est une estimation, et non une cartographie précise, la population couverte présentant, de plus, quelques biais et lacunes. Élargir la couverture du territoire est donc une nécessité, et la création d'un registre général à l'échelon national y contribuerait. Cette proposition de loi répond à une forte demande, exprimée par de nombreuses institutions depuis plusieurs années. Ainsi, les commissions d'enquête sénatoriales sur les risques industriels et sur la pollution des sols, en 2020, ont formulé des conclusions en ce sens. L'Igas a souligné, la même année, que des données à échelle géographique plus fine sont nécessaires, particulièrement lors de repérages de clusters à des fins de recherche et de santé publique. nationale de médecine, dans son rapport de 2021, appelle à la création d'un registre national des cancers, afin de collecter les données épidémiologiques et d'assurer progressivement un enregistrement national des cancers géographiquement représentatif. L'objet de ce registre national serait, sur la base des registres existants, de centraliser les données et de recenser les cas de cancers de façon exhaustive sur l'ensemble du territoire national, mais aussi de constituer un outil de veille sanitaire et d'alerte épidémiologique. L'INCa en serait l'hébergeur et le gestionnaire administratif, le réseau Francim des registres des cancers pourrait assurer les aspects techniques et scientifiques, l'évaluation des données et leur analyse. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement européen de création et d'harmonisation des registres des cancers, la couverture de l'ensemble de la population étant déjà disponible dans 22 pays européens

pour la surveillance de l'incidence du cancer et de la mortalité par cancer dans l'Union européenne. Cette base de données à l'échelle de l'Europe constitue une source précieuse, pouvant être exploitée à des fins de recherche, sur la base d'un protocole établi par les équipes scientifiques et validé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le champ des recherches est vaste : l'épidémiologie, les facteurs de risques éventuels, la qualité des soins, l'efficacité des traitements, les conséquences environnementales sur les cancers, dont l'importance croissante mérite une veille accrue. Il comprend également l'évaluation de déterminants géographiques et sociaux, qui pourraient être à l'origine de politiques et d'actions de réduction des inégalités en matière de santé que nous connaissons à l'heure actuelle.

Il frappe sans discernement, quels que soient notre âge, notre sexe ou notre origine. Selon les données de l'OMS, le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, avec des millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année. En France, avec 382 000 nouveaux cas et 157 000 décès annuels, le cancer est la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. Ces chiffres sont alarmants, mais ils ne doivent pas nous décourager. Au contraire, ils doivent nous inciter à agir et à développer des stratégies, afin de lutter contre cette terrible maladie. C'est pourquoi le RDSE salue l'initiative de notre collègue, le docteur Sonia de La Provôté, ainsi que le travail de notre rapporteure, Nadia Sollogoub. Le texte que nous examinons aujourd'hui entend en effet donner les outils nécessaires pour mettre en place des stratégies plus efficaces de prévention, de dépistage et de diagnostic. La surveillance épidémiologique des pathologies cancéreuses repose sur l'enregistrement et le suivi continu et exhaustif des nouveaux cas de cancer grâce aux registres qui ont été créés progressivement depuis les années 1970. Mais la couverture du territoire reste partielle, puisque l'on ne dénombre que 33 registres et que les registres généraux non spécialisés ne couvrent que 22 % de la population française. La mise en place d'un registre national est une demande récurrente depuis plusieurs années. Le Conseil scientifique international estimait en Le Conseil scientifique international estimait en 2020 que l'INCa devrait jouer « un rôle de leader dans la création de ressources nationales pour le partage et l'intégration des données, le soutien et la recherche en matière de nouvelles initiatives thématiques. Plus récemment, l'Académie nationale de médecine a appelé à la création d'un registre national des cancers, afin d'accélérer les remontées d'informations nécessaires à l'exercice d'une mission de surveillance sanitaire élargie. La mise en place d'un tel outil marquerait par ailleurs une étape importante en vue d'une prochaine harmonisation européenne. Rappelons qu'un nombre croissant de nos voisins, tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Suède, se sont dotés de registres ayant une couverture nationale. Mes chers collègues, je le répète, la centralisation des données relatives aux cancers sur l'ensemble du territoire national est nécessaire pour améliorer la prévention et le dépistage, dont le rôle est essentiel pour lutter contre cette maladie et sauver des vies. Une étude lancée au mois de février 2021, l'étude Cascade, dont l'objectif est de dépister le cancer du poumon grâce à un scanner à faible dose, chez les femmes, en France, vient de livrer ses premiers résultats une participante sur trente a été dépistée positive. Il en ressort qu'à consommation de tabac égale, les femmes seraient plus exposées que les hommes au risque de développer cette maladie. Alors qu'il baisse nettement chez les hommes, le cancer du poumon continue de monter de façon exponentielle chez la femme tend à devenir la première cause de mortalité par cancer, devant celui du sein. Cette étude relance l'idée d'un dépistage systématique des fumeurs. Souvent diagnostiqué à un stade tardif, le cancer du poumon de plus mauvais pronostic et celui qui occasionne le plus de décès. Un dépistage organisé permettrait d'agir de manière proactive et de détecter les cas de cancer du poumon à un stade précoce lorsque les chances de guérison sont les plus élevées. Pour toutes les raisons

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avec 380 000 nouveaux cas diagnostiqués par an, le cancer reste la première cause de mortalité prématurée en France. un ennemi à combattre ! Depuis les années 1970, il existe des registres généraux ou spécialisés qui permettent une surveillance épidémiologique des cancers. Pour rappel, un registre est une structure qui réalise « un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une équipe ayant les compétences appropriées Les registres des cancers sont un dispositif indispensable à la surveillance des cancers, mais aussi à l'observation et à l'évaluation de leur prise en charge. Ils permettent de connaître, globalement et selon les organes concernés, le nombre et le taux de cancers, la durée de survie, et l'évolution de ces paramètres dans le temps. Les données populationnelles recueillies dans ces registres contribuent à l'orientation, au suivi et à l'évaluation des politiques de santé publique dans le domaine de la lutte contre les cancers. Elles participent également aux actions préventives et curatives, ainsi qu'à la recherche. Ces registres sont nécessaires au suivi épidémiologique et à la programmation des besoins en structures de soins. Il est vrai que la couverture des registres de cancers permet déjà de disposer de chiffres robustes. Le dispositif national s'appuie sur les données de 33 registres, qui couvrent environ 22 % de la population française métropolitaine et trois départements et régions d'outre-mer. Pour les enfants, le registre national des cancers de l'enfant est exhaustif sur l'ensemble du territoire national depuis 2011. La surveillance des cancers repose actuellement sur un dispositif qui est piloté par l'Institut national du cancer et Santé publique France, en partenariat avec les registres des cancers fédérés au sein du réseau Francim et le service de biostatistique et bio-informatique des Hospices civils de Lyon. Ce partenariat prévoit la publication d'estimations nationales d'incidence et de survie tous les cinq ans. La collecte des données épidémiologiques du cancer en France a fait de réels progrès grâce aux efforts des registres régionaux et départementaux. Cependant, la couverture du territoire reste partielle, et il existe une hétérogénéité des structures et des modalités de recueil des données. les difficultés financières sont réelles et le rendu des données est lent, avec la production d'un rapport tous les cinq ans seulement. La récupération de données est, en effet, complexe. Elle demande du temps et un financement non négligeable. L'enregistrement des données doit être exhaustif et précis, et l'utilisation de celles-ci doit respecter la loi Informatique et libertés, avec notamment une obligation de sécurité. Il ne faudrait pas que la complexité du recueil et du traitement des données au niveau national constitue un obstacle dirimant à la mise en place d'un registre national des cancers. Malgré l'évidente utilité des registres existants, le dispositif présente certaines limites, qui nous interrogent sur l'efficience du modèle actuel, notamment l'exhaustivité du recueil des données et leur financement. Par ailleurs, l'absence d'une stratégie nationale et d'une coordination entre les registres fragilise l'utilisation de ces données, avec la production d'un rapport tous les cinq ans seulement. C'est pourquoi je suis favorable à la création d'un registre national des cancers. De nombreux pays, comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, réalisent déjà des compilations à l'échelle nationale, ce qui leur permet de mieux comprendre et prendre en charge les cancers. Dès 1995, l'Allemagne a légiféré sur l'obligation, pour les seize états fédérés, de mettre en place des registres épidémiologiques des cancers, afin de bénéficier d'un registre national. Ces registres contiennent des données importantes, du diagnostic à l'issue de la maladie, en passant par les traitements et les récidives. Je tiens à souligner que la création du registre national s'est accompagnée de financements importants. Le budget alloué à la mise en place des registres cliniques des cancers est de 7,2 millions d'euros. Il est financé par la ligue allemande contre le cancer. Les frais courants des registres s'élèvent à 140 euros par cas et sont pris en charge à 90 % par les caisses d'assurance maladie et à 10 % par les. Le Le coût d'un registre est donc important. En France, pour les registres des cancers, qui couvrent environ 20 % de la population, 8 millions d'euros sont dépensés chaque année pour le seul recueil des cas, auxquels viennent s'ajouter les coûts d'exploitation des données et des études portant sur ces données. La création d'un registre national des cancers doit donc impérativement être accompagnée d'un financement à la hauteur des enjeux de santé publique qu'il représente. Nous attendons du Gouvernement qu'il s'engage à la soutenir financièrement. ailleurs, ce registre national pourrait être articulé avec d'autres sources de données, par exemple des données d'exposition, ce qui pourrait permettre l'identification d'associations entre exposition et survenue de cancer. À titre d'exemple, la Suède a ainsi pu établir très tôt un lien entre le tabagisme au cours de la grossesse et le cancer de l'enfant. Le registre national des cancers permettra de couvrir l'ensemble du territoire et de procéder à l'enregistrement continu de toutes les données permettant la production d'un rapport annuel.

Ce texte ajoute aux missions de l'INCa la « mise en oeuvre d'un registre national des cancers », qui centralisera les données relatives aux cancers sur l'ensemble du territoire national, afin d'améliorer la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des malades du cancer, mais aussi de constituer un outil de suivi et d'alerte épidémiologique, ainsi qu'une base de données à des fins de recherche. Le rapatriement des données du registre à l'INCa facilitera leur appariement avec celles du système national des données de santé, auxquelles l'Institut a un accès permanent. Ce texte complète également les missions de l'INCa, en l'autorisant à labelliser des entités de recherche en cancérologie, afin d'encourager la constitution d'équipes de collecte de données, et l'habilite à développer et à héberger des systèmes d'information dans les domaines de la cancérologie, afin de faciliter l'hébergement des données des registres existants existants par l'Institut, dont la solution technique est sûre et souveraine. La mise en place de ce registre national des cancers sera un outil supplémentaire et précieux dans la lutte contre cette maladie. Pour être réellement efficace, l'outil aura besoin de financements. La parole

En 2018, on dénombrait 382 000 cas de nouveaux cancers. L'incidence de certains types de cancers, comme ceux du foie, du poumon ou du pancréas, ne cesse d'augmenter. Et, depuis les années 1990, partout dans le monde, le nombre de personnes de moins de 50 ans atteintes d'un cancer ne cesse de croître. Ainsi, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant, grâce à cette proposition de loi, que la France ne disposait pas d'un registre national des cancers Je ne suis ni médecin ni chercheur, et j'étais persuadée qu'un tel outil existait déjà dans notre pays. Sa création est pourtant l'objet de la proposition de loi de notre collègue Sonia de La Provôté, qui préconise de mettre en place un registre qui centraliserait les données relatives aux cancers sur l'ensemble du territoire. Cette idée mérite considération. Il existe déjà une vingtaine de registres qui couvrent différents départements, et une douzaine d'autres, spécialisés et ciblés sur le recensement de certains types de cancers. Mais ces registres ne couvrent au final que 24 % de la population. Le calcul de l'incidence et de la prévalence à l'échelon national se fait donc avec des estimations, qui, aussi utiles qu'elles puissent être, n'en restent pas moins des extrapolations. La collecte de données de ce type représente un véritable travail de fourmi, qui nécessite de croiser de nombreuses sources : celles des hôpitaux, des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'imagerie médicale ou encore celles de l'assurance maladie. Même si les méthodes ont fait beaucoup de progrès, différentes études ont montré que les modes de recueil des données varient entre les registres existants. Il peut en résulter un manque d'exhaustivité ou des doublons. En outre, la restitution reste lente, le rendu se faisant tous les cinq ans. Des extrapolations ne peuvent pas tenir compte, à mon sens, des spécificités et des facteurs propres à un territoire, d'autant plus quand certains liens de cause à effet sont encore méconnus. En 2010, par exemple, des manifestants ont envahi l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) et réclamé les chiffres du nombre de cancers à Fos-sur-Mer et, plus largement, autour de l'étang de Berre, site particulièrement industrialisé. Certains habitants pensaient qu'on leur cachait des choses, mais le fait est que ces chiffres étaient tout simplement indisponibles, car il n'existait pas de registre pour cette zone. Autre exemple : un article que j'ai lu il y a peu disait qu'environ 100 000 nouveaux cas de cancers de la peau sont dépistés chaque année en France. Ce chiffre double tous les dix ans. En 2022, on comptait même 150 000 nouveaux cas. Cet article indiquait également que les départements de Loire-Atlantique et de Vendée étaient les plus touchés. Or ces deux territoires sont justement dotés chacun d'un registre des cancers. Si un tel outil existait pour chaque département, cela ne permettrait-il pas de comparer les données, d'expliquer potentiellement les causes d'une surincidence, voire de découvrir de nouveaux facteurs de risque ? Nous pensons que l'instauration d'un registre couvrant l'intégralité du territoire national représenterait une véritable avancée. Certes, tous les acteurs ne soutiennent pas cette initiative, les responsables de l'INCa au premier chef, mais leur argument tient surtout à la question du coût d'une telle mesure, sans qu'ils remettent en question son intérêt. À notre sens, l'argument financier, s'il compte évidemment, ne peut pas prévaloir quand on parle d'un outil qui permettrait de fournir un maximum de données pour améliorer la recherche, la prévention, le dépistage et le traitement de l'une des premières causes de mortalité chez nos concitoyens.

le papyrus chirurgical, rédigé dans l'ancien système d'écriture égyptien, contenait déjà, vers 1 500 avant notre ère, une référence à un cancer du sein. Il appartient, au même titre que les archives médicales, aux sources indirectes. Aujourd'hui, les registres constituent un outil épidémiologique précieux pour les

-ou sur des sites sensibles. À la suite des petits pays scandinaves et de l'Allemagne, nous devons tendre vers un registre national populationnel pour une meilleure analyse des expositions aux facteurs de risque environnementaux et socioprofessionnels. De plus, il convient d'harmoniser les systèmes informatiques, d'homogénéiser les données et de pérenniser, comme cela a été dit, le financement sans perte d'énergie pour boucler les budgets. Le registre national permettra de publier chaque année, et non tous les cinq ans, l'incidence des cancers, la consommation de soins nous renseignant quant à elles sur leur prévalence. Le registre national populationnel répondra aux demandes des associations de dépister rapidement les foyers de surincidence de certains cancers, les nouveaux et les signaux faibles, en lien avec de possibles facteurs environnementaux. Enfin, avec ce registre national, la France bonifiera sa contribution au réseau européen des registres des cancers, notamment pour les cancers rares.

Par exemple, des études démontrent que, chez les femmes, le travail de nuit augmente de 26 % le risque de cancer du sein. De leur côté, des chercheurs suédois ont mis en avant le risque que présente le travail féminin impliquant une manipulation de papier journal.

de la maîtrise des dépenses de santé se trouve dans la politique de prévention. Or celle-ci sortira renforcée de ce dispositif, alors que les coûts des traitements des cancers explosent

améliorer le dépistage, la prévention, le traitement et le suivi des cancers. C'est en effet indispensable. Toutefois, il existe depuis 1975 des registres nationaux, qui couvrent une partie du territoire.

loi que nous examinons aujourd'hui, présentée par notre collègue Sonia de La Provôté, a pour but de créer un registre national des cancers. Ce registre centralisera les données populationnelles relatives à l'épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie sur l'ensemble du territoire. Le traitement de ces données sera confié à l'Institut national du cancer. Ce registre permettra notamment de connaître le nombre exact de cancers et les foyers de surincidence et ainsi d'orienter l'offre de soins, la prise en charge thérapeutique et, bien sûr, les politiques de prévention.

Ce registre constitue donc un outil épidémiologique au service d'une plus grande efficacité de la prise en charge des cancers en France, mais aussi, bien sûr, une base de données pour alimenter les travaux de recherche. La création d'un tel registre s'inscrit également dans un mouvement européen d'harmonisation, car il viendrait alimenter le réseau européen des registres du cancer. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain partage bien évidemment les objectifs de cette proposition de loi.

couvrent, de manière inégale, entre 22 % et 24 % de la population nationale. De plus, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), ces données présentent des caractéristiques particulières qui freinent leur croisement avec d'autres, en particulier celles du SNDS ou celles des certificats

L'Agence européenne pour l'environnement estime que les risques d'origine environnementale ou professionnelle sont responsables d'environ 10 % des cancers. De la même manière, en France, on estime à 40 % le taux de cancers qui pourraient être évités par le développement d'environnements et de comportements favorables. Il paraît donc primordial d'intégrer dans ce nouveau registre national des données environnementales afin de permettre la mise en oeuvre de politiques publiques, en particulier de politiques publiques de prévention.

réhabilitation de ces sols. Dans ce dernier rapport, Gisèle Jourda estimait que les registres des cancers pourraient être ouverts pour mieux évaluer le lien entre l'apparition de certains cancers et l'exposition, par exemple, à l'arsenic dans l'Aude ou à des métaux lourds dans le Gard- ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'apparition de cancers des poumons. Le groupe SER souhaite donc que l'une des missions du registre national des cancers soit d'évaluer les conséquences sur la santé humaine de l'exposition à des substances polluantes.

porté essentiellement par l'INCa et Santé publique France, est stable depuis plus de dix ans, alors que le nombre de cancers ne cesse d'augmenter. De plus, le décompte des cas de cancer en France requiert des ressources humaines. Or qui dit ressources humaines dit financement. Il apparaît que les registres sont alimentés médicale (Inserm), par des équipes d'accueil universitaires ou encore par des associations qui supportent elles-mêmes, en propre, le coût de cette collecte. Madame la ministre, il n'est pas dans nos prérogatives de parlementaires d'agir sur cet aspect financier. Je m'adresse donc à vous pour que,

sur des travaux récents de l'Académie de médecine, vise à mettre en place un registre national des cancers. C'est un sujet qui lui tient à coeur, comme elle l'a souligné. Je veux également remercier la rapporteure, Nadia Sollogoub. En France, les cancers demeurent la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme. Les cancers les plus fréquents diagnostiqués pour les femmes sont le cancer du sein- 33 %-et pour les hommes le cancer de la prostate- 24,6 %. Les inégalités socio-économiques pèsent lourd dans la mortalité liée au cancer. si cette maladie peut toucher tout le monde, elle frappe plus durement les personnes les moins éduquées. Une étude du Centre international de recherche sur le cancer, menée dans dix-huit pays européens, confirme à quel point la position socio-économique augmente le risque de mourir de cette maladie. Ce n'est pas surprenant, quand on sait que la prévention des cancers repose essentiellement sur le dépistage auquel les gens recourent inégalement Ainsi, dans le cas du cancer du col de l'utérus, 75 % des femmes les plus modestes de 25 à 34 ans ont recours au dépistage contre 87 % des plus aisées, tandis que, pour le cancer du sein, 61 % des des femmes les plus modestes de 50 à 74 ans ont recours au dépistage contre 76 % chez les plus aisées. Enfin, les cancers d'origine professionnelle demeurent sous-estimés, alors même que près de 10 % des salariés en France sont exposés à un ou plusieurs agents cancérogènes au cours de leur activité professionnelle. Chez les ouvrières et les ouvriers, la part des cancers imputables à l'activité professionnelle atteindrait près de 20 %. Ce résultat est sans doute sous-estimé, car, jusqu'à présent, la recherche de l'origine professionnelle d'un cancer se heurte à une traçabilité incomplète des expositions au cours de l'exercice de l'activité professionnelle. Dans la plupart des cas, attribuer l'origine d'un cancer à des causes professionnelles relève d'un travail d'investigation complexe qui nécessite de pouvoir retracer l'historique des expositions de chaque salarié. Dès lors, la proposition de ce texte de créer un registre national pour centraliser les données relatives aux cancers de l'enfant et de l'adulte sur l'ensemble du territoire national nous paraît tout à fait pertinente. Cet outil épidémiologique permettra de fournir des données populationnelles populationnelles précieuses pour l'observation des cancers et l'orientation des politiques de santé publique, mais également pour alimenter les travaux de recherche. Il s'agit, par conséquent, d'une contribution précieuse à l'amélioration de la connaissance et donc de la prévision des cancers. Ce registre national sera un atout pour évaluer les actions préventives et curatives menées et pour détecter l'évolution des facteurs de risque. Il est regrettable que le Comité national des registres créé en 1996 ait été supprimé en 2013 et que les trente-trois registres des cancers territoriaux ou spécialisés ne couvrent que 22 % de la population générale. Nous espérons que ce retard sera rattrapé, en confiant à l'INCa la gestion du registre national ; nous espérons surtout, madame la ministre, que l'État apportera son soutien financier à ce dispositif afin de ne pas créer de nouvelles déceptions.

ou (PALB 2)- pour n'en citer que quelques-unes. Pour les personnes porteuses de ces mutations, le risque de souffrir d'un cancer au cours de leur vie est donc plus élevé que dans la population générale. Le registre national des cancers proposé par la présente proposition de loi a pour objet d'améliorer la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des cancers. De ce fait, il paraît opportun de collecter également les données relatives aux prédispositions génétiques aux cancers, puisque la détection d'anomalies génétiques participe à la prévention et nécessite la mise en place de dépistages réguliers. En outre, la prise en charge thérapeutique peut être adaptée en cas de mutation génétique et la collecte de telles données peut être utile pour la recherche. Le présent amendement vise donc à préciser que le registre national des cancers centralise également les données relatives aux anomalies génétiques prédisposant aux cancers, y compris lorsqu'un cancer n'est pas déclaré. Quel est l'avis de la commission ? Le registre

Pour vous en convaincre, permettez-moi de porter la voix d'habitants de mon département, situés dans la plaine d'Aunis, à proximité de La Rochelle. Là, entre 2009 et 2018, six enfants au moins ont développé des cancers. L'histoire est connue, la presse nationale l'a relatée à plusieurs reprises- encore hier, dans l'hebdomadaire, dont je vous recommande la lecture. Concrètement, qu'est-ce qui a permis aux médecins des familles concernées de vérifier leur constat empirique de cas anormalement concentrés de cancers ? Qu'est-ce qui a permis d'objectiver la situation pour agir ? Eh bien, vous n'en serez pas surprise, il s'agit de l'existence d'un registre des cancers. Sans cela, un temps précieux aurait été perdu. Ce registre a montré combien il était nécessaire dans le cas d'espèce. Est-il suffisant pour autant ? Loin de là ! Depuis qu'il a permis de partager le constat, le chemin restant à parcourir pour établir les causalités et déterminer les facteurs de risque sociaux et environnementaux est long et laborieux. les parents et citoyens de la plaine d'Aunis font preuve d'un esprit de responsabilité et d'un sang-froid remarquables. L'agglomération de La Rochelle joue avec volontarisme un rôle qui- cela me coûte de le dire -devrait être celui de l'État, qui rase les murs sur le sujet. C'est l'agglomération qui organise des réunions publiques, qui commande des campagnes de mesures de qualité de l'air, qui demande à ses agents de consacrer du temps pour faire se parler les acteurs de terrain- familles, élus, médecins, entreprises, agriculteurs, associations, etc. Je voulais donc saisir l'occasion de ce débat pour vous demander, madame la ministre, de passer un message à votre excellent collègue ministre de l'agriculture. Il s'était engagé à nous transmettre, pour septembre 2022, une étude de l'Agence toujours repoussée depuis lors sans aucune explication- y compris à l'adresse des journalistes qui l'interrogent. Cela devient indécent et ne peut entraîner que de la suspicion. Or, pour éviter la suspicion- c'est notre sujet -et pour permettre un débat constructif, rien de mieux que des données ouvertes et accessibles. Les difficultés pour établir les causalités et les prises de conscience sur les cadres sociaux et environnementaux favorisant les cancers suffisent à justifier que nous ne privions pas 75 % du territoire national de cette première étape indispensable de caractérisation des foyers de cancer, comme nous en avons bénéficié en Charente-Maritime. C'est donc avec conviction que je voterai avec mon groupe cette proposition de loi.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Union Centriste, de la proposition de loi relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic, présentée par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues (proposition

le contrôle aérien est un service public essentiel pour notre pays. Il participe de notre souveraineté, permet d'assurer le contrôle de notre espace aérien et assure un rôle majeur pour nos territoires et pour la connectivité du pays, un rôle régalien.

aujourd'hui que ce service public est engagé dans une modernisation qui lui permet de rejoindre le peloton de tête européen dans le cadre du « ciel unique » et de l'interopérabilité.

navigation aérienne, que nous avons le devoir de trouver une solution qui soit conforme à nos traditions. Il convient bien sûr de respecter le droit de grève : c'est le pilier de cette proposition de loi. C'est bien parce qu'existe

J'ai essayé de proposer une solution à un problème ancien. Je souhaite le faire dans le cadre du dialogue social. Je veux aussi dire combien je suis attaché à la modernisation de cette belle maison qu'est la DGAC. Tout cela ne peut passer

relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic. Ce texte porte sur un sujet bien identifié par le grand public : les conséquences sur le trafic aérien des mouvements sociaux des contrôleurs aériens employés au sein de la direction générale de l'aviation civile. Le cadre Le cadre actuel de ces mouvements sociaux n'est pas satisfaisant. Certes, les organisations syndicales de la DGAC doivent déposer un préavis de grève cinq jours avant le début de tout mouvement, mais il est très difficile pour l'administration d'anticiper l'ampleur réelle de chaque La DGAC n'a actuellement aucun moyen de savoir avec précision combien d'agents décideront d'y participer. Il résulte de cette situation d'incertitude que les abattements de vols fréquemment bien plus élevés que nécessaire, afin d'éviter les annulations de dernière minute, dites « à chaud », qui sont les plus pénalisantes pour les compagnies aériennes comme pour les passagers. La réduction du trafic qui résulte de la grève est donc disproportionnée au regard de la participation parfois très faible du personnel au mouvement. Le fonctionnement actuel est déroutant : il permet aux contrôleurs aériens d'annoncer qu'ils vont faire grève sans avoir besoin de réellement passer à l'action. Comme les « abattements » de vols ont lieu avant avant le début du mouvement, les effets recherchés de la grève sur la réduction de trafic sont déjà atteints avant même qu'elle ne commence. parfois, que la DGAC ait une analyse trop optimiste de la situation et annule en amont moins de vols qu'il n'aurait été nécessaire. Il faut alors procéder en urgence à des annulations « à chaud Celles-ci désorganisent très fortement le trafic aérien. Des passagers déjà arrivés dans les terminaux, voire dans les avions, voient leur vol annulé. Cela peut donner lieu à des troubles à l'ordre public, liés à la présence dans les aéroports de nombreuses personnes courroucées face à ces situations difficiles. Cette incertitude est en outre pénalisante pour les contrôleurs aériens eux-mêmes. En cas de grève, il est en effet possible de déclencher un dispositif de service minimum, afin d'assurer la continuité du service public et une certaine partie des opérations, en particulier celles liées aux vols vers la Corse et les outre-mer et au survol du territoire français. La DGAC est donc souvent obligée de déclencher préventivement ce dispositif, et ce même quand le nombre de grévistes s'avère en définitive faible, si bien qu'il n'aurait pas été nécessaire de le mettre en place. Ce service minimum implique des réquisitions de personnel. Les contrôleurs réquisitionnés ne peuvent,, participer au mouvement de grève, quand bien même ils l'auraient voulu. Le service minimum a aussi pour effet de fragiliser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Parfois, le service minimum peut même être mis en place assez tardivement. Il est alors difficile de notifier aux contrôleurs leur réquisition et il arrive- dans de rares cas, il est vrai -que les forces de l'ordre doivent s'en charger. Cette situation n'est évidemment pas pleinement satisfaisante. Au cours des derniers mois, ce système a montré ses limites de façon très claire, en particulier le 11 février dernier, quand des contrôleurs aériens ont rejoint une grève de la fonction publique qui n'avait même pas été relayée en interne par les syndicats de la DGAC. Il en a résulté de nombreuses annulations à chaud. Les semaines suivantes, le service minimum a été fréquemment mis en place, ce qui a dégradé le climat de travail à la DGAC, ce dispositif étant lourd de conséquences et complexe à organiser tant pour les contrôleurs aériens que pour leur direction. La coupe du monde de rugby et les jeux Olympiques approchant à grands pas, une réforme de ce système est plus que jamais nécessaire. La présente proposition de loi vise à remédier à cette situation. Elle crée une obligation, pour les contrôleurs aériens, de se déclarer individuellement grévistes l'avant-veille du mouvement de grève, avant midi. Ils ont la possibilité de renoncer à leur participation au mouvement jusqu'à dix-huit heures le même jour. Sur la base de ces informations, l'autorité administrative pourra décider de mettre en place le service minimum. Elle disposera, pour ce faire, d'un délai contraint : également jusqu'à dix-huit heures l'avant-veille du mouvement. L'information contenue dans les déclarations permettra à l'autorité administrative de déterminer avec précision le nombre de vols à annuler. Les adaptations du trafic aérien seront donc mieux proportionnées à l'ampleur du mouvement, et les annulations à chaud pourront ainsi, nous Cette déclaration individuelle s'inscrirait dans le prolongement de déclarations similaires existant déjà dans le secteur des transports, depuis 2007 dans le transport terrestre régulier de voyageurs et depuis 2012 pour les autres travailleurs du secteur aérien. Les contrôleurs aériens n'avaient pas été inclus dans le champ de la loi Diard de 2012 créant une obligation de déclaration individuelle de participation à la grève, car ce texte ne concernait que le secteur privé,

En commission, nous avons adopté un amendement tendant à préciser qu'elles seront couvertes par le secret professionnel. En outre, toute utilisation à d'autres fins que celles prévues dans le texte serait passible de sanctions pénales. La proposition de loi reprend donc le principe de la loi Diard, mais n'en constitue pas un simple calque. En effet, il était notamment nécessaire de veiller ici à l'articulation entre la déclaration individuelle et le service minimum. Pour l'examen de cette proposition de loi, j'ai cherché à m'inscrire dans une philosophie de recherche de l'équilibre et de pragmatisme. Le texte adopté par la commission est pleinement en phase avec cette exigence. Il est adapté au cadre d'exercice des contrôleurs aériens et remédie à ses principales insuffisances. Il crée certes une obligation pour les contrôleurs, la déclaration individuelle, mais il en crée également une pour l'administration, puisque le délai de déclenchement du service minimum est contraint. Le texte résorbe les principales difficultés du système actuel pour les passagers, puisque moins de vols seront annulés préventivement et « à chaud », mais aussi pour les contrôleurs aériens, puisque le service minimum sera déclenché moins souvent

Ce déclenchement, nécessaire pour assurer, conformément à la loi, la continuité du service public essentiel de la navigation aérienne, se décide en effet sur la base d'éléments d'information partiels, épars et parfois subjectifs. Pour éviter de devoir annuler des vols « à chaud », ce qui est le plus pénalisant pour les usagers

Ce texte rend ainsi obligatoire l'envoi d'une déclaration individuelle de participation au mouvement de grève, au plus tard à midi l'avant-veille d'une journée de grève, pour les agents des services de la navigation aérienne qui assument

et les contrôleurs pourront exercer effectivement leur droit de grève sans être systématiquement astreints. Nous aurons ainsi un meilleur service et un exercice garanti et plus efficace du droit de grève.

Le Gouvernement est donc, vous l'aurez compris, favorable à cette proposition de loi qui, je l'espère, saura recueillir une large majorité des suffrages dans cet hémicycle. Bien sûr, le dialogue devra continuer avec l'ensemble des parties prenantes pour assurer une mise en oeuvre de ce texte qui soit en adéquation avec les besoins de chacun et les grands principes que j'ai rappelés.

par l'entreprise ou le secteur concerné. Par ailleurs, il s'agit toujours d'une forme de gestion de la pénurie, le droit de grève restant d'ordre constitutionnel. On a encore pu le constater « à chaud » en ce début d'année avec les contestations massives de la réforme des retraites. Je salue l'initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas, ancien maire du Bourget, qui vise à apporter une réponse à un problème bien connu des usagers du transport aérien. Je rappellerai ici l'engagement de notre ancienne collègue et membre du groupe RDSE, Josiane Costes, en faveur des lignes d'aménagement du territoire, les LAT. En 2019, elle avait signé un rapport d'information sur la contribution du transport aérien au désenclavement et à la cohésion des territoires, en particulier de ceux qu'il faut bien appeler de véritables « îles intérieures », comme son département du Cantal. Dans nos fonctions de parlementaires, nous sommes souvent confrontés à des perturbations, retards ou annulations de vols, alors que les moyens de transport alternatifs n'existent pas toujours, ou en tout cas pas avec le même temps de transport. Et je ne vous dis pas ce qu'on entend sur les contrôleurs aériens dans les avions ou les aéroports ministre, qu'en est-il de la stratégie nationale du transport aérien 2025 ? A-t-elle porté ses fruits ? Quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui, à mi-parcours, et alors que Paris accueillera en 2024 les jeux Olympiques, exactement un siècle après leur première organisation dans la capitale ? D'après le rapport sur la présente proposition de loi, entre 2004 et 2016, deux tiers des grèves du contrôle aérien en Europe ont eu lieu en France. Les clichés semblent ainsi, hélas, se vérifier, avec un impact certain sur le trafic en Europe, compte tenu de la situation géographique de notre pays. L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est l'un des trois ou quatre premiers aéroports du continent en nombre de passagers annuels. Il serait intéressant de connaître l'évolution depuis 2016. La situation actuelle se caractérise par un dévoiement des dispositifs liés au droit de grève, dans un sens comme dans l'autre, avec une déconnexion croissante entre l'ampleur d'une grève et son impact sur le trafic, du fait des annulations préventives par la DGAC et du déclenchement du service minimum par précaution, pour pallier le manque d'information. Face à cette situation, les réquisitions semblent elles-mêmes montrer leurs limites. Il s'agit donc bien d'un problème d'organisation et d'anticipation, auquel cette proposition de loi vise à répondre. Mme la rapporteure défend même l'idée que ce texte contribuerait paradoxalement à renforcer le droit de grève, en le faisant mieux appliquer dans les faits.

aux déclarations individuelles de participation à une grève : cela contribue à protéger le droit de grève, qui est, rappelons-le, d'ordre constitutionnel. En conclusion, les membres du groupe RDSE devraient se prononcer pour l'adoption de cette proposition de loi, à l'exception de quelques abstentions.

Face à ce constat implacable, la proposition de loi de notre collègue Vincent Capo-Canellas est plus que nécessaire. Aujourd'hui, la DGAC ne connaît pas à l'avance le nombre de contrôleurs participant à une grève, car ces derniers sont exemptés de se déclarer grévistes avant la grève elle-même. Le système de prévention et d'information actuellement en place a largement démontré sa totale inadaptation à la réalité des opérations. Comment expliquer qu'aujourd'hui, en France, les contrôleurs aériens n'aient aucune obligation de prévenir leur direction de leur participation à une grève alors qu'ils doivent assurer un service minimum comme celui prévu pour le transport terrestre de voyageurs ou pour d'autres métiers du secteur aérien ? Comment expliquer que, faute de prévisibilité, la DGAC annule préventivement des vols ou procède à des annulations de dernière minute, laissant les clients sans solution ?

-qui confondent tour de contrôle et tour d'ivoire ! Oui, le métier de contrôleur- comme d'autres métiers, d'ailleurs -est un métier à haute responsabilité ; ceux qui l'exercent doivent gérer une multitude d'informations pour assurer la sécurité des passagers.

adapter les demandes de réduction de programme à la réalité du suivi du mouvement et donc éviter des annulations inutiles ou des attentes interminables.

Le service minimum et le respect des voyageurs ont la même valeur pour tous, que ce soit en train, en bus ou en avion. Il faut atterrir, mes chers collègues ! Le service minimum, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Il ne s'agit certainement pas de solder de vieilles querelles.

Je souhaite que le Sénat et le Gouvernement restent mobilisés sur le sujet, car de nombreux défis doivent encore être relevés pour sortir du mythe actuel et organiser enfin un véritable service minimum. que cette proposition de loi ne s'attaque pas aux préavis de grèves dormants, dont tout un chacun peut se réclamer, alors qu'ils datent parfois de plusieurs années. Je déplore également que l'on ne puisse pas aller plus loin, en allongeant le délai de déclaration individuelle de grève, pour avoir encore plus de lisibilité. Toutefois, cette proposition de loi constituant un début de réponse non négligeable à une situation devenue intolérable, le groupe Les Républicains la votera sans réserve. Très bien ! La

préserver le droit de grève, constitutionnel, tout en garantissant la continuité du service public aérien, qui est essentiel à la vie économique et sociale de la Nation. L'attractivité et la fiabilité des aéroports français sont directement concernées. Nous avons travaillé pour trouver un équilibre entre l'ampleur du mouvement social et la baisse du trafic. Cela passe par une meilleure anticipation et plus de prévisibilité, tout en préservant le droit de grève. Je salue le travail effectué en commission par notre collègue rapporteure Évelyne Perrot. L'objectif démocratique de cette proposition de loi étant largement partagé dans cet hémicycle, faisons évoluer cet outil pour le rendre plus efficace, à la fois

le déclenchement du service minimum par précaution n'est pas une situation satisfaisante pour les différents acteurs en présence. Disposer d'une vision sur le contingent réel des contrôleurs aériens grévistes afin d'organiser le trafic aérien national et international relève du bon sens. Or seule l'anticipation le permet.

Mes chers collègues, vous l'avez compris, le groupe Les Indépendants est attaché au droit de grève et à son exercice par les contrôleurs aériens, dès lors que les répercussions sont proportionnées. Les contrôleurs aériens ne peuvent pas être plus longtemps exonérés des règles qui régissent le droit de grève. les usagers ne méconnaissent pas le rôle essentiel des contrôleurs aériens dans l'organisation et la sécurité du trafic, ils estiment que, dans une société moderne comme la nôtre, ils doivent pouvoir s'organiser en amont, lorsque la profession fait valoir son droit de grève. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants

le sujet qui nous occupe est éminemment sensible, dans la mesure où il touche à des libertés aussi essentielles que celles de se déplacer ou de faire grève. En tant que fonctionnaires, les contrôleurs aériens ne peuvent participer à une grève que s'ils sont couverts par un préavis de cinq jours francs.

aériens doivent assurer un service minimum depuis la loi de 1984 et son décret d'application avec un taux de réquisition variable. Il leur est ainsi

façon- disons-le ! -, une réaction aux perturbations qu'a provoquées en février et mars derniers l'exceptionnelle et puissante mobilisation populaire contre la retraite à 64 ans. connu un 11 février sans service minimum, puis un mois et demi avec un service minimum quasi permanent, mais souvent disproportionné, aux dépens des voyageurs. Pour autant- disons-le aussi ! -,

qui assurent les fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte, lorsque leur absence est de nature à empêcher des vols. Ce dispositif me paraît clair, ciblé,

de commandement, des services administratifs aux usagers. Cette transmission d'une information fiable permettra une meilleure organisation et une adaptation

le débat n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre l'avion. Le secteur aérien participe de l'avenir de la mobilité durable.

Les graves perturbations du trafic aérien ces derniers mois, avec quarante jours de grève entre la mi-février et la fin mars, marqueront l'année 2023. La journée mémorable du 11 février- la

Permettez-moi, monsieur le ministre, de m'interroger sur la façon dont la DGAC a géré la situation. En l'état, il est clair que l'application du service minimum avec réquisition de contrôleurs aériens n'a pas permis de gérer la situation de manière optimale.

Il est indispensable de rediscuter et de réactualiser les obligations du service minimum afin de le rendre plus efficace. Actuellement, l'application du service minimum est à géométrie variable. est totale sur la manière dont sont opérés les « abattages » de vol. Si le décret d'application précise la liste des aéroports où ce service minimum peut être appliqué et les missions de continuité

j'estime qu'il est urgent de renouer le dialogue social et de retrouver la confiance entre les agents et la direction, car l'année 2023 a fortement altéré la démocratie sociale au sein de la profession. Les contrôleurs aériens sont des fonctionnaires qui assurent des missions hautement stratégiques,

Il est temps que le Gouvernement agisse ! Si nous adoptons ce texte, deux types d'obligations et de contraintes pèseront sur les contrôleurs aériens, sans pour autant avoir réformé le service minimum. Les agents favorables à la proposition de loi souhaitent que cette nouvelle obligation de déclaration préalable individuelle de grève soit conditionnée à une diminution des obligations de service minimum.

Madame la présidente, monsieur le ministre,

échu d'avoir à assurer la pérennité des activités civiles de cinq aéroports entre mars 2007 et septembre 2020. Ces treize années, en toute modestie, m'ont permis de vivre un petit échantillonnage des turbulences économiques et sociales qui secouent le monde du transport aérien.

pour illustrer le fait que la catégorie professionnelle dont il est question s'occupe aussi d'autre chose que du décollage ou de l'atterrissage des avions sur un aéroport donné

Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour le secteur aérien. Comme l'a très justement rappelé la rapporteure, Évelyne Perrot, le déroulement des grèves consécutives à la réforme des retraites au sein de la direction générale de l'aviation civile a montré de façon très claire les limites du système actuel. Il n'y a aucune prévisibilité du trafic : la DGAC doit naviguer- ou plutôt piloter -à vue pour déterminer la proportion de vols à annuler, car elle ne dispose d'aucun outil pour connaître suffisamment tôt le nombre de contrôleurs aériens qui participeront à un mouvement de grève. Quelques grévistes peuvent conduire à des abattements massifs de vols et engendrer de fortes perturbations, en totale disproportion avec l'ampleur réelle du mouvement. Le double objectif de cette proposition de loi est donc tout à fait louable

Des dispositifs analogues existent déjà pour tous les autres professionnels du secteur aérien, ainsi que dans le secteur ferroviaire, et ils ont fait la preuve de leur efficacité.

elle met simplement un terme à une aberration : le fait que des grèves très peu suivies, souvent déclenchées pour des motifs complètement extérieurs au transport aérien, perturbent fortement le trafic.

Ces derniers ont tout à gagner à ce qu'il soit adopté, afin que le service minimum soit organisé avec plus de sérénité et, surtout, que l'on y recoure moins fréquemment. Le dialogue social en sortira très renforcé.

Les compagnies françaises sont les plus touchées par les conséquences des grèves du contrôle aérien. La proportion de vols qu'elles ont assurés en mars dernier par rapport à mars 2019 n'est que de 85 %, contre 88 % pour les compagnies étrangères. elles doivent faire face à de très nombreux défis pour mener à bien la transition écologique et elles font preuve d'un engagement intense pour décarboner leur activité. Dans ce ciel incertain, il est nécessaire de limiter au maximum les turbulences que rencontre le secteur, afin qu'il retrouve sa vitesse de croisière le plus rapidement possible. Je soutiens donc pleinement l'excellente initiative de Vincent Capo-Canellas, qui a su mener un exercice de haute voltige : écrire un texte qui soit acceptable pour tous et qui résolve, avec le moins de contraintes possible, un maximum de situations problématiques. Je l'en remercie, ainsi que la rapporteure, Évelyne Perrot, qui s'est pleinement investie sur ce sujet aussi complexe qu'essentiel pour nos concitoyens. La parole

et que nous partirions au moins avec une heure de retard- « quand les aiguilleurs du ciel l'auront décidé », nous a indiqué le pilote. Affolement dans l'avion pour tous ceux qui, comme moi, avaient une correspondance.

Malgré ses insuffisances, seize ans après, je constate qu'elle a pu améliorer la prévisibilité des perturbations sans empêcher le droit de grève- on nous reprochait à l'époque

Cela a été rappelé, le droit de grève des aiguilleurs du ciel remonte à bientôt quarante ans. La réquisition alors prévue, qui devait permettre d'assurer 50 % des arrivées et des départs, n'a pas fonctionné.

Entre les grèves que font les contrôleurs du ciel pour leurs conditions de travail, celles qu'ils font pour des conditions locales, celles qu'ils font en tant que fonctionnaires contre la réforme des retraites, et sans doute pour bien d'autres raisons que nous ignorons, que ce texte changera quelque chose ! Monsieur le ministre, je comptais vous demander si vous seriez celui qui oserait enfin appliquer une disposition qui n'a rien d'excessif.

Il y a quelques années, quatre compagnies aériennes européennes ont déposé une plainte contre la France, le survol de l'Hexagone leur ayant été interdit pour près de seize mille vols en un seul trimestre. ou, qui regroupe seize compagnies réclame cette année à la Commission européenne d'imposer une protection des survols en cas de grève, mesure qui existe déjà en Italie. Monsieur le ministre, allez-vous agir vite et éviter une condamnation de la France ? Pouvez-vous confirmer aussi que, pour éviter les zones de contrôle aérien français, les transporteurs ont volé en moyenne 96 000 kilomètres de plus par jour de grève, ainsi que l'indique Eurocontrol

rapporteur engagé sur ces questions.

concertée de travail par au moins deux agents de l'autorité administrative concernée. En effet, cela ne va pas vous surprendre, les préavis de grève illimités rendent les anticipations impossibles. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement a

notamment dans le code des transports. En effet, la loi du 16 janvier 1984 prévoit que « l'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation

permettrait au personnel gréviste de renoncer à la grève, non pas vingt-quatre heures avant chaque journée de grève, comme le prévoit la loi Diard, mais la veille de la journée, à dix-huit heures. Cette situation laisserait trop peu de temps à l'autorité administrative pour réaliser les « abattements » de vol et, le cas échéant, organiser le service minimum, ce qui va à rebours de l'objectif de la les contrôleurs aériens ne bénéficieraient pas non plus de l'organisation plus en amont du service minimum que vise à mettre en place le texte que De surcroît, aucune mesure de coordination entre ce nouveau délai et celui qui est laissé à l'administration pour déclencher le service minimum, lequel resterait l'avant-veille à

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chaque année, nous finissons par évoquer la question de l'ouverture du mécénat aux sociétés publiques locales (SPL) culturelles. Nous poursuivons ainsi la tradition- la série, devrais-je plutôt dire -, après les saisons 2019, 2020, 2021 et 2022, marquées par le dépôt d'amendements à des projets de loi de finances ou dans le cadre de lois relatives aux collectivités territoriales, par exemple la loi L'ouverture du mécénat aux SPL culturelles est donc devenue un cheval de bataille sénatorial. Constante dans ses votes, notre assemblée a toujours soutenu, à l'unanimité, cette mesure. À certains moments, nous n'étions pas loin qu'elle devienne réalité, mais les compromis issus des commissions mixtes paritaires lui ont été systématiquement défavorables, charriant regrets et déceptions. C'est pourquoi, en cette saison 2023, nous avons décidé d'innover et de « taper plus fort », afin d'inverser le cours de cette histoire. Ainsi, c'est par le biais d'une plus par voie d'amendement, que nous voulons permettre aux SPL culturelles de bénéficier du mécénat. J'utilise à dessein le pronom « nous », car il faut souligner qu'il s'agit d'une initiative transpartisane, traduisant fidèlement l'esprit de concorde qui unit le Sénat sur ce sujet. Les temps de concorde étant actuellement rares, savourons-les. J'espère que le Gouvernement, faisant preuve de la sagesse qui le caractérise, s'y joindra avec entrain. En cette occasion, je salue et associe pleinement mes collègues Julien Bargeton, Hervé Marseille et Antoine Lefèvre, coauteurs de cette proposition de loi et partenaires précieux dans ce combat en faveur des collectivités territoriales et de la décentralisation. En effet, cette proposition de loi vise avant tout à développer la culture et l'attractivité des territoires, en revenant sur une inégalité de traitement flagrante entre l'État et les collectivités. Rappelons que, à la lecture de l'article 238 du code général des impôts, impôts, l'État, « [seul] ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales », peut recourir au mécénat afin de financer des projets culturels. L'État et les collectivités territoriales peuvent donc s'associer et faire appel au mécénat pour mettre en place de tels projets. de loi consacre ainsi cette logique d'association, vertueuse et si caractéristique de l'exercice de la compétence culturelle partagée, en l'appliquant aux collectivités territoriales qui s'unissent et qui désirent recourir au mécénat en vue de la réalisation d'un projet culturel. En d'autres termes, il ne s'agit nullement de créer un dispositif, dérogatoire au droit commun et spécifique aux collectivités, il s'agit bien plutôt de leur permettre ce que l'État s'autorise. En ce sens, ce texte répare une inégalité- d'aucuns diraient même une injustice. Objectivement, quel argument pourrait justifier cette rupture d'égalité entre l'État et les collectivités, alors même que le périmètre du mécénat, ainsi que les finalités visées sont strictement identiques ? Est-ce à dire que les collectivités territoriales seraient moins légitimes à s'associer entre elles pour développer des projets culturels le mécénat ? Est-ce à dire que les collectivités territoriales seraient moins garantes de l'intérêt général ? Est-ce à dire que les collectivités territoriales seraient moins précautionneuses quant aux conditions de recours au mécénat ? Je ne le crois absolument pas et, comme vous vous en doutez, monsieur le ministre, le Sénat ne pourrait que s'inscrire en faux devant une telle défiance. En effet, il ne s'agit que de confiance. Le Gouvernement est-il enfin prêt à faire confiance aux collectivités regroupées sous forme de SPL qui voudraient déployer une ambition culturelle sur leur territoire ? Quand il est question de décentralisation, souvent sont invoqués un territorial, un acte III, y compris d'ailleurs au sein du Gouvernement, mais la décentralisation peut aussi être approfondie par la méthode des petits pas, chère à Robert Schuman et Jean Monnet. Ce texte est un tout petit pas décentralisateur. Si vous n'êtes pas décidé à y consentir, comment pourrions-nous croire en la détermination réelle du Gouvernement de « mener ensemble une nouvelle étape pour une vraie décentralisation » ? Saisissez donc cette proposition de loi comme un moyen de prouver en actes la confiance que vous revendiquez d'accorder aux collectivités. Par ailleurs, j'ai entendu les questionnements juridiques que pouvait faire naître ce texte. J'aimerais y apporter plusieurs réponses. Premièrement, en vertu de l'article L. 1531-1 général des collectivités territoriales, les seuls actionnaires des SPL sont les collectivités territoriales. Cet actionnariat public permet aux collectivités d'oeuvrer en commun pour mener des actions d'intérêt général. Mutualisation, souplesse, partenariat public-public à l'échelle locale et subsidiarité effective peuvent ainsi caractériser ces entreprises publiques locales (EPL). Deuxièmement, les SPL ne peuvent pas créer de filiale et se contentent d'agir pour le compte de leurs collectivités actionnaires. Troisièmement, en aval, les SPL font l'objet de contrôles multiples et renforcés. S'il était besoin de rassurer, nous pourrions même affirmer qu'elles sont les structures les plus contrôlées ! Elles le sont par les

tant en interne qu'en externe, ce qui apporte de nombreuses garanties. Quatrièmement, la loi 3DS et ses décrets d'application ont affermi les règles en matière de déontologie, de transparence et de prévention des conflits d'intérêts applicables aux EPL.

culturelles ou patrimoniales, par analogie au régime qui prévaut pour les dons et legs faits aux communes. Par conséquent, l'édifice visant à prévenir les conflits d'intérêts est consolidé, pour ne pas dire parachevé. Du point de vue budgétaire, vue budgétaire, des réticences ont été exprimées. Soyons précis : nous parlons d'une dépense fiscale estimée à 1,7 million d'euros par an, par an, laquelle ne prend aucunement en compte les retombées fiscales et économiques indirectes qu'elle génère : augmentation des recettes de la TVA et des taxes de séjour, ainsi que de l'emploi et de l'activité économique dans les territoires concernés. Lors des auditions que j'ai menées, tous mes interlocuteurs, du MuséoParc Alésia au Palais des papes d'Avignon, ont insisté sur cet aspect : la culture sert de levier pour renforcer l'attractivité touristique et économique des territoires. L'ouverture du mécénat aux SPL élargirait la palette aux mains des collectivités pour dynamiser leur territoire. Les incertitudes étant aujourd'hui nombreuses, il devient fondamental d'octroyer un maximum de moyens aux collectivités, tout en les laissant libres d'y recourir. C'est pourquoi je ne pourrai pas comprendre un quelconque dogmatisme qui s'arrêterait à l'évidence, considérant qu'il s'agit d'une dépense fiscale. Oui, et alors ? A-t-elle une incidence positive sur l'activité ? Oui ! Rapporte-t-elle aux collectivités, ainsi qu'à l'État ? Oui ! La dépense fiscale n'est pas mauvaise en soi, si elle est un investissement, ce qui est le cas. J'ajoute qu'une évaluation du dispositif sera toujours possible- elle sera même souhaitable et bénéfique -, afin de mesurer ses effets aussi bien sur les finances publiques que sur l'activité économique, les collectivités territoriales

Parallèlement, d'autres inquiétudes ont émergé eu égard à la dégradation très nette de l'environnement global. Je pense au renchérissement du coût de l'énergie, mais pas seulement. Pour le dire clairement, les arts et la culture sont fragilisés dans les discussions budgétaires, terrain de prédilection du résurgent combat idéologique et civilisationnel, comme on le voit aujourd'hui. Il faudra probablement ouvrir une réflexion pour rendre la compétence culture obligatoire et rénover la matrice de nos politiques publiques

écot à cet objectif. Elle fait partie d'une politique plus large de sauvegarde, de développement et de valorisation de la vie culturelle de nos territoires. Répondant à la fois à un besoin et à un désir de mécénat de proximité, elle conduirait également les collectivités à amplifier leur politique culturelle, le recours au mécénat n'étant ouvert aux SPL que si leur activité principale est de nature culturelle. Élan décentralisateur, rigueur juridique, en particulier dans le contrôle, dépense faible par rapport au retour sur investissement, instrument au service d'une ambition et d'une vision culturelle du territoire, les raisons sont multiples et variées de soutenir cette initiative. Connaissant l'attachement du Sénat à cette mesure, je ne doute pas de son soutien plein et entier ; en revanche, j'espère sincèrement que le Gouvernement s'y montrera favorable et qu'il enverra ainsi un signal positif à la fois

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France est un pays connu à travers le monde pour son rayonnement culturel,

permet d'animer et d'essaimer l'action culturelle sur l'ensemble du territoire national. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

il y a vingt ans, la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Aillagon, donnait un nouvel élan au mécénat en France, en permettant que les versements des entreprises au bénéfice d'organismes dont l'objet est culturel, philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial ouvrent droit à une réduction d'impôt. Aujourd'hui, un ensemble de trois réductions d'impôt est ouvert aux entreprises et aux particuliers au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière. L'effet de levier fiscal recherché par la loi Aillagon est devenu la colonne vertébrale du soutien à la générosité dans notre pays. Pour nos finances publiques, cela représente chaque année un effort important de plus de 3 milliards d'euros près de 1,1 milliard d'euros pour le mécénat des entreprises, 1,8 milliard d'euros pour les dons des particuliers et plus de 130 millions d'euros au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Ce système permet à chaque donateur de choisir, parmi un large éventail d'activités d'intérêt général,

des activités des organismes qui diffusent notre culture, notre langue et nos connaissances scientifiques ; des activités d'aide à la création d'entreprises ; enfin, des activités à caractère sportif et culturel, ainsi que de celles des organismes qui mettent en valeur notre patrimoine artistique ou organisent des spectacles. Le champ culturel, objet de la présente proposition de loi, est particulièrement bien couvert. Les arts plastiques, la musique, la danse, le théâtre et les spectacles, le livre et la littérature, le cinéma et l'audiovisuel, le patrimoine et la connaissance du patrimoine, les musées, le développement de la vie culturelle, la formation artistique, le dialogue entre les cultures, les liens entre la vie culturelle et la vie économique ou scientifique ou encore la restauration des monuments : toutes ces activités sont aujourd'hui éligibles au dispositif d'exonération fiscale. Le mécénat permet aussi la prise en compte de contributions en nature, comme le mécénat de compétences des entreprises ou encore certains frais engagés par les bénévoles au profit des associations dont ils sont adhérents. Ce soutien fiscal s'accompagne enfin d'autres exonérations, notamment en matière de donation. Je pense en particulier à l'exonération de droits de donation pour les dons au profit des organismes éligibles à la réduction d'impôt sur la fortune immobilière, qui représente environ 100 millions d'euros chaque année. C'est donc un dispositif très complet qui laisse à chaque Français et à chaque entreprise une grande liberté pour choisir celles des causes d'intérêt général qu'il souhaite voir l'État soutenir financièrement. Cette liberté de choix, c'est la clé du succès du dispositif de la loi Aillagon. Cet environnement fiscal, nous devons le préserver pour ses vertus. C'est pour cela que cette majorité a souhaité, en 2020, relever le plafond de versements pour les petites entreprises, en portant ce montant de 10 000 euros à 20 000 euros. C'est aussi pour cela que des aménagements temporaires ont été prévus pour de grandes causes nationales, comme la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la suite du tragique incendie de l'année 2019, ou pour lutter contre les violences domestiques. Pendant la crise sanitaire, nous avons également relevé le taux applicable aux dons aux associations caritatives venant en aide aux plus démunis. Nous avons aussi, avec le prélèvement à la source, introduit une amélioration considérable, en intégrant la réduction d'impôt pour les particuliers dans le champ de l'avance versée en janvier : chaque année, désormais, les foyers qui ont effectué des dons éligibles au titre de l'avant-dernière année se voient verser à cette date Nous avons enfin aménagé le régime de TVA des dons des entreprises et introduit des dispositions favorables pour les entreprises qui donnent des biens achetés dans le cadre de leur activité économique à certaines associations. Vous le voyez, le Gouvernement a considérablement mobilisé le levier fiscal au service de cette nécessaire générosité. Préserver le mécénat, c'est aussi se garder de toute dérive et rester fidèle aux grands principes qui le rendent légitime pour les Français, qui, à travers leurs impôts, contribuent à soutenir les dons éligibles à ces différentes formes de soutien fiscal.

la rémunération des dirigeants de l'entité. Enfin, les organismes soutenus ne doivent pas être lucratifs. Cela signifie en particulier qu'ils ne peuvent pas prendre la forme d'une société commerciale. C'est l'un des points au coeur de la discussion. Je sais le Sénat particulièrement sensible à la bonne utilisation des deniers publics. C'est pourquoi le Gouvernement, ces dernières années, a travaillé avec votre assemblée, et le Parlement en général, au renforcement du dispositif de contrôle de la défiscalisation des dons. Cette Cette sensibilité est partagée, entre autres, par la Cour des comptes. Comme vous le savez, dans son rapport de novembre 2018, la Cour insistait sur le dynamisme de la dépense fiscale, notamment pour les entreprises, dans un contexte marqué par la baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés.

Elle prévoit de le faire dans deux situations précises : lorsque ces sociétés ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque

En premier lieu, nous devons à tout prix éviter, dans les incitations fiscales à la générosité, d'organiser une hiérarchie des causes d'intérêt général. Je pense que nous ne serions pas collectivement en mesure d'expliquer pourquoi les activités que je viens de citer seraient éligibles à un dispositif dans une situation où les versements au profit d'associations caritatives,

pour objet d'étendre très substantiellement une disposition, elle-même dérogatoire, mais circonscrite. Les termes actuels de la loi garantissent que cette exception reste minimale par une condition forte : la présence de l'État au capital. Le Gouvernement est d'avis que cette exception doit être préservée. Ouvrir des dérogations supplémentaires pourrait fragiliser la cohérence d'ensemble de ce que le législateur définit comme une activité non lucrative et d'intérêt général. En troisième lieu, le volet de votre proposition de loi relatif au patrimoine aboutit à intégrer dans le champ de la réduction d'impôt, uniquement lorsque ces activités sont exercées par des sociétés lucratives, des activités qui ne sont aujourd'hui même pas éligibles à la réduction d'impôt de droit commun. La rédaction vise ainsi l'accès à tous les biens immobiliers et mobiliers qui présentent un intérêt esthétique ou encore les pratiques sociales et les événements festifs. Elle va au-delà de la notion de patrimoine retenue aujourd'hui pour l'application du régime du mécénat.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le mécénat culturel est un moyen à la fois ancien et efficace de soutenir toutes les formes de création artistique et la préservation de notre patrimoine.

efficace, dans la mesure où il constitue une alternative au soutien public : on l'a vu lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, qui a suscité un afflux exceptionnel de promesses de dons, souvent défiscalisées il est vrai, ou encore avec le loto du patrimoine, qui a rencontré un réel engouement depuis sa mise en place. Le secteur culturel et surtout, sans surprise, le spectacle vivant ont été fortement touchés par les restrictions liées à la crise sanitaire, bien qu'ils aient aussi bénéficié des largesses du « quoi qu'il en coûte ». Le mécénat culturel est aujourd'hui principalement le fait des entreprises, grandes ou moins grandes, mais il dépend fortement de la conjoncture et de la santé économique desdites entreprises, qui auront tendance à réduire en premier ce poste de dépenses en cas de difficultés.

l'exercice de la compétence culture étant partagé avec l'État. La volonté de trouver de nouvelles sources de financement est louable et rappelle des discussions que nous avions déjà eues il y a deux ans

On peut aussi penser à la réserve parlementaire, supprimée en 2017, qui était un levier d'investissement dans le patrimoine local en dépit des défauts qui ont conduit à sa disparition. La présente proposition de loi étend un avantage fiscal octroyé aux TPE et PME qui font du mécénat culturel aux dons en faveur des sociétés publiques locales détenues par des collectivités, indépendamment de la participation ou non de l'État. Elle a été déposée par des sénateurs issus des

seulement une cinquantaine de structures en France : les sociétés publiques locales à vocation culturelle. Nous ne sommes pas naïfs, les entreprises trouvent aussi un avantage à s'engager dans le mécénat culturel, car elles bénéficient ainsi de retombées en termes d'image de marque et de visibilité locale, en plus de l'avantage fiscal lui-même. La semaine dernière, la commission des finances a adopté des précisions de nature à garantir un meilleur suivi de l'usage de ces fonds et à éviter les conflits d'intérêts au sein des SPL. On sait que c'est une préoccupation très

par la loi du 28 mai 2010, les sociétés publiques locales ont confirmé le rôle déterminant qu'elles jouent dans l'exécution de missions d'intérêt général au service des collectivités. En complément de leurs prérogatives en matière d'aménagement et de gestion des services publics industriels et commerciaux, c'est dans le domaine de la culture que leur intervention a démontré son intérêt majeur. Elles ont ainsi pu contribuer à renforcer l'action de l'État, notamment lors de la crise sanitaire, les longs mois de fermeture administrative ayant lourdement pénalisé les métiers de la culture et du spectacle vivant.

Les exemples ne manquent pas : des établissements culturels, connus et reconnus, comme la tour Eiffel, le Palais des papes à Avignon, le château des ducs de Bretagne à Rennes ou encore l'abbaye royale de Fontevraud dans le Maine-et-Loire, sont administrés sont administrés et financés par des collectivités réunies en société publique locale. À ces sites renommés s'ajoute toute une liste de théâtres, musées, cinémas, festivals ou centres culturels, répartis sur l'ensemble du territoire et dont le modèle de gestion et de contrôle a fait la preuve Ouvrir aux sociétés publiques locales le mécénat culturel et le régime fiscal qui y est associé apparaît ainsi comme un moyen de reconnaître à leur juste valeur leur action en faveur de la culture, de favoriser l'investissement dans des établissements « à domicile » et ainsi, de participer au rayonnement culturel de la France et de ses territoires. Le dispositif incitatif que ce texte propose de créer se substitue ainsi aux investissements dans des établissements implantés à l'étranger, qui offrent sinon un régime de mécénat plus avantageux. De plus, la gouvernance des sociétés publiques locales étant intégralement publique, elle procède directement des décisions adoptées par les collectivités représentées au sein de leur conseil d'administration. La relation interne qui en résulte permet non seulement de déroger aux contraintes des règles de mise en concurrence prévues dans le code de la commande publique, mais elle assure de surcroît un contrôle direct sur les actions de la société publique locale. La loi 3DS du 21 février 2022 a renforcé par ailleurs les règles de ce contrôle, en prévenant les risques de conflit d'intérêts et en associant les chambres régionales et territoriales des comptes et les commissaires aux comptes à l'obligation de suivi de leur activité. La société publique locale étant sans but lucratif, sa gestion désintéressée la protège contre les risques de malversation,

des sociétés publiques locales dépasse les sensibilités politiques. J'espère que l'Assemblée nationale sera sensible à ce travail transpartisan dans l'intérêt de nos territoires et pour la vitalité de la culture à la française.

Grand. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le monde de la culture a été durement éprouvé par la pandémie. Pour de très nombreux acteurs, les mesures sanitaires ont remis en cause l'essence même de leur activité. Qu'est-ce qu'un théâtre, qu'est-ce qu'un cinéma, qu'est-ce qu'un musée sans public ? La culture a payé un lourd tribut à la lutte contre le virus. Au-delà de l'épreuve humaine, la pandémie a également durement éprouvé les modèles économiques des acteurs de la culture. Ils ont été privés de ressources et la dynamique de création, qui suppose l'échange, a été mise à mal. Bien sûr, le Gouvernement et le Parlement se sont très tôt mobilisés pour soutenir tous ces acteurs, notamment ceux de nos territoires, qui, partout en France, font vivre la création à chaque coin de rue- des associations et des collectivités sont ainsi mobilisées.

nous ouvrons de nouveaux modes de financement à ces acteurs des territoires et nous créons des liens avec les entreprises. L'initiative est d'autant plus forte qu'elle est transpartisane. Je précise qu'elle aurait été encore plus forte si elle avait été omnipartisane ... Notre groupe la soutiendra néanmoins.

Nous souhaitions mobiliser davantage de fonds privés au bénéfice des SPL.

Désormais, la consommation des biens culturels passe aussi par les nouvelles technologies. Dès lors, il apparaît nécessaire d'adapter notre cadre législatif à cette nouvelle donne. Il est important d'adopter les codes de la jeunesse pour faciliter son accès à la culture.

Le propos de notre collègue Sylvie Robert sur le volet décentralisateur est limpide et je le partage entièrement. Malgré le soutien massif des pouvoirs publics, la pandémie a fortement affecté le secteur de la culture. Le spectacle vivant retrouve difficilement son public. L'inflation a pour effet d'accroître plus encore la baisse de réduire la mixité des publics. Ainsi, 70 % des médiathèques et des bibliothèques n'ont pas retrouvé la fréquentation antérieure à la pandémie. Les métiers techniques sont en tension. De nombreux artistes et auteurs n'arrivent plus à faire face à la triple précarité- contrats courts, pluriactivité, bas salaires -qui caractérise les emplois du secteur, comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport de mai 2022.

D'après les travaux du Conseil économique, social et environnemental, la situation ne va pas s'améliorer, puisque les directions des affaires culturelles annoncent, dans leurs notes de cadrage budgétaire,

début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. [ ...] « Il faut qu'ils sachent que, ô merveille, ils ont une oeuvre, faite de mille oeuvres, à accomplir, ensemble [ ...]. « Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la genèse n'est pas encore terminée et qu'elle leur appartient ?

À ce jour, l'article 238 du code général des impôts dispose que seuls les dons destinés à certains organismes d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Les dons en faveur des musées de France et d'organismes culturels dont l'un des actionnaires est l'État ou des établissements publics nationaux entrent ainsi dans ce cadre. Par ce biais, les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des dons dans la plupart des cas, et à 40 % pour les dons qui excèdent 2 millions d'euros. L'abaissement du taux ne concerne cependant pas les dons faits au profit d'organismes à but non lucratif venant en aide aux personnes en difficulté en facilitant leur accès au logement ou en leur fournissant gratuitement un repas, des soins, voire des produits produits de première nécessité. Concernant le sujet qui nous occupe, le rapporteur, que je remercie pour la qualité de son travail, a largement répondu aux arguments qui avaient jusqu'à présent justifié la suppression du dispositif à l'Assemblée nationale. J'ai souhaité les reprendre ici, car ils sont déterminants pour notre position sur ce texte. L'une des alternatives proposées à l'élargissement des dons aux sociétés publiques locales consiste à créer un fonds de dotation ou un établissement public en association avec l'État. Pour autant, cela ne répondrait pas correctement à la question du financement : les dons destinés aux SPL seraient soumis à la TVA et la création d'un établissement public engendrerait des coûts de fonctionnement importants. À l'inverse, les SPL, en contribuant à un partenariat entre plusieurs acteurs publics, conduiraient à une rationalisation des ressources.

et Michel Canévet, notre rapporteur, pour cette proposition de loi, qui coûtera peu à l'État, mais éclairera l'action culturelle dans nos collectivités territoriales. Sur cette base, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. La

Nous avons donc besoin d'innover pour relancer le secteur. La proposition de loi de notre collègue Sylvie Robert, dont je salue l'engagement actif et de longue date en faveur de la culture, est de nature à apporter un nouvel outil aux collectivités territoriales pour faciliter les investissements en la matière.

L'exercice partagé de la compétence culture avec l'État favorise une dynamique qui permet le développement de projets culturels à l'échelle locale. Cependant, lorsque les conjonctures économiques deviennent défavorables, le risque de désengagement cumulatif est très fort.

En ouvrant le mécénat culturel aux SPL à vocation culturelle ou patrimoniale, nous envoyons un signal de confiance fort à l'ensemble des élus territoriaux, qui nous semblent être les mieux à même de construire des politiques culturelles de proximité répondant aux attentes de leurs concitoyens.

Concrètement, le dispositif proposé fait converger le souhait des collectivités territoriales d'une plus grande souplesse dans leur action culturelle et la volonté d'engagement des entreprises au niveau local.

La question du coût pour nos finances publiques est également bien maîtrisée : environ 1,7 million d'euros, soit moins de 1 % des 230 millions d'euros que représente le mécénat culturel chaque année.

pour éviter le risque de conflits d'intérêts. Notre groupe votera donc en faveur de ce texte et souhaite son adoption par nos collègues de l'Assemblée nationale afin qu'il entre en vigueur dans les meilleurs délais.

hauteur de 2,85 millions d'euros à cette forme d'action publique culturelle. À ce jour, notre territoire ne compte que 51 sociétés publiques locales à vocation culturelle, dont une seule dans mon département du Nord. Contrairement aux crédits budgétaires, qui garantissent une péréquation de l'offre culturelle,

La culture est un domaine dans lequel les collectivités territoriales sont pleinement investies, y compris financièrement. Elles fournissent près de 70 % de l'investissement public en faveur du secteur culturel en France, soit un montant annuel de 9,5 par an, les SPL à vocation culturelle, dont elles détiennent l'intégralité du capital et déterminent les missions. Cependant, cet effort financier consacré à un secteur vital pour l'attractivité des territoires est aujourd'hui menacé les coûts additionnels engendrés par la crise sanitaire et, plus récemment, la hausse des coûts de l'énergie ont fragilisé la situation budgétaire des collectivités et en particulier leur capacité d'investissement.

face auxquelles la France accuse un retard significatif. Alors que la dette de notre pays atteint des niveaux sans précédent, il serait regrettable de faire reposer sur les acteurs publics, et plus encore sur les collectivités territoriales, le coût des investissements nécessaires au redressement du secteur culturel.

ils ne sont pas suffisamment attractifs pour les acteurs privés que sont les TPE, les PME et les ETI présentes dans les territoires. Ces dernières redirigent donc leurs efforts vers des acteurs privés ou vers des sociétés publiques dont l'État est lui-même actionnaire. que l'État puisse mobiliser le mécénat culturel alors que les collectivités territoriales, qui contribuent le plus au financement du secteur culturel, ne le peuvent pas ? Ce texte permettra de remédier à cette injustice et offrira au secteur culturel de nouvelles sources de financement, tout en soulageant les collectivités d'un fardeau

Les sociétés chargées de l'accès du public au patrimoine, qui participent au rayonnement de nos territoires, pourront également en bénéficier. Cela déclenchera à l'évidence un appel d'air en faveur du financement privé des initiatives des collectivités en matière culturelle, d'autant plus que la culture et la préservation du patrimoine sont le deuxième domaine d'action privilégié des entreprises, après le sport, et que 80 % des entreprises mécènes engagées dans le secteur culturel le sont au niveau local. Afin de prévenir tout risque de conflits d'intérêts, la commission a prévu que les dons devront être autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés publiques locales. Ce dispositif offre ainsi toutes les garanties de sécurité juridique nécessaires à un financement transparent et utile du secteur culturel. Au vu de ces considérations,

ces dernières doivent-elles assumer seules cette responsabilité ? Absolument pas. Qu'il s'agisse d'investissements économiques ou de culture, le dynamisme de nos territoires passe par l'essor et l'encouragement des initiatives privées. d'autant plus vrai que le mécénat, dont vous avez détaillé la composition, monsieur le rapporteur, concerne avant tout les petites entreprises, soit celles qui font la richesse d'une région par les emplois qu'elles y créent et par l'attachement réciproque qui se noue entre un territoire et ses acteurs économiques. Si des entreprises sont désireuses de consacrer une part de la valeur qu'elles ont créée à la culture locale, ne boudons pas notre plaisir ! Il me semble donc nécessaire de faire sauter certains verrous juridiques qui brident inutilement les initiatives. Cette ouverture encadrée du mécénat en faveur des sociétés publiques locales permettra notamment de financer la mise en valeur de notre patrimoine, car l'attachement que nous lui portons n'a d'égal que le coût de sa restauration. Châteaux, petites églises non classées, maisons de caractère, ce bâti est le socle de l'identité culturelle de nos communes et sa préservation exige la participation de tous les acteurs de la société : l'État,

Je soutiens donc pleinement ce texte, lequel réaffirme une volonté maintes fois exprimée par le Sénat, et notamment par les rapporteurs de la loi 3DS, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud. Darnaud. Incitons les entreprises à enrichir, par leurs dons, le capital culturel de leur territoire, favorisons l'émergence des Jacques Coeur, Peggy Guggenheim ou Pierre Cardin du XXI siècle, car, plus que jamais, le rayonnement culturel sera, demain, un facteur de prospérité

Cette initiative audacieuse, portée en particulier par Colette Mélot et ses collègues du groupe Les Indépendants - République et Territoires, mérite d'être saluée et encouragée. Cette proposition de loi intervient à un moment crucial de notre histoire, où l'art numérique connaît une expansion sans précédent. Les médias et les experts en parlent comme d'une véritable révolution culturelle. Un terrain d'expression artistique se dessine dans lequel la créativité rencontre les avancées technologiques ; cela nous rappelle que l'art est capable de s'adapter aux progrès de notre société. Grâce à la démocratisation des outils numériques et à la facilité d'accès à internet, l'art numérique peut désormais toucher un large public, transcendant les frontières géographiques et les barrières sociales, générationnelles et culturelles. L'article 1 de cette proposition de loi revêt une importance particulière : il vise à intégrer l'art numérique dans le champ du mécénat. Cette mesure incitera les particuliers et les entreprises à soutenir financièrement les réalisations artistiques numériques. à l'esprit les spectacles son et lumière organisés dans nos villages et dans nos villes, qui sont l'occasion de valoriser notre patrimoine et nos monuments historiques, de promouvoir notre héritage culturel et de contribuer au développement économique et touristique de nos territoires.